La séance est suspendue. La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réformer l'adoption n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. En conséquence, l'examen de ses conclusions, initialement inscrites, sous réserve de leur dépôt, jeudi 16 décembre prochain, est retiré de l'ordre du jour du Sénat.

Madame la présidente,

de jours de congé de présence parentale (CPP), c'est-à-dire à ceux qui s'occupent d'un enfant malade, victime d'un accident ou en situation de handicap. Le nombre maximum de jours de CPP et d'AJPP dont peuvent bénéficier des parents pour un enfant est fixé à 310 jours dans la limite d'une durée de trois ; ce droit à 310 jours de CPP et d'AJPP peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie, après que la période de trois ans est écoulée. Dans les faits, 95 % des situations sont traitées par ce dispositif. Un approfondissement était cependant nécessaire. C'est bien l'objet de ce texte, que le Gouvernement soutient pleinement. Un trou dans la raquette de la loi du 8 mars 2019 faisait que le droit au renouvellement de l'AJPP ne pouvait être rouvert qu'après l'expiration du délai de trois ans. Cela ne permettait pas de répondre aux situations caractérisées par des traitements longs, nécessitant un arrêt total d'activité de la part de l'un des parents, et ce sur une période très prolongée. Cela ne concerne que les 5 % des bénéficiaires de l'AJPP qui vont jusqu'au bout des 310 jours, soit

également prévu de permettre, à titre exceptionnel et par dérogation au dispositif actuel, de renouveler une fois la période de trois ans sans attendre la fin du terme de la première période de trois ans et d'ouvrir ainsi droit à un nouveau compteur maximal de 310 jours de CPP et d'AJPP, dans la limite des trois années à venir,

je crois savoir qu'il reçoit l'approbation de l'ensemble des groupes politiques, je tiens à revenir sur quelques points afférents qui, eux aussi, ont un impact sur le quotidien des parents d'enfants malades. Il y a tout d'abord la question, souvent relevée, des complexités administratives que le circuit de traitement des demandes de CPP et d'AJPP n'est pas encore optimal. Sachez à ce propos, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'il est prévu de mieux croiser les fichiers et d'aller vers une récupération automatique de la plupart des ressources des bénéficiaires, afin de simplifier les démarches les démarches des allocataires et de favoriser le juste recours aux prestations. Ainsi seront utilisées les données issues des flux de la déclaration sociale nominative liées à la déclaration de la suspension du contrat de travail pour le motif d'octroi d'un congé de présence parentale. La comptabilisation du nombre de jours de congé pris par le salarié permettra aux organismes de suivre directement les situations et d'effectuer les versements dans des délais beaucoup plus courts.

J'évoque ce point, car il s'agit justement de l'un des attendus de la mission que le Gouvernement vient de confier au député Paul Christophe. Vous le savez sans doute, le travail collectif engagé sur l'accompagnement des parents d'enfants malades ne s'arrêtera pas avec la promulgation du texte dont nous discutons aujourd'hui- bien au contraire ! M. Christophe aura pour mission, au cours des prochains mois, de dresser le panorama le plus large possible de ces questions, d'identifier précisément les publics concernés, de cibler les manques et les faiblesses des dispositifs existants et de proposer le cas échéant des améliorations de notre système.

de formation des travailleurs sociaux et d'accompagnement psychologique. C'est véritablement un sujet auquel le Gouvernement attache beaucoup d'importance. Les travaux de M. Christophe permettront, j'en suis convaincu, d'améliorer le traitement des dossiers et, par conséquent, l'accompagnement des parents au quotidien.

proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Adoptée par l'Assemblée nationale voilà près d'un an, elle est très attendue des associations, qui espèrent une entrée en vigueur rapide de ses dispositions. Créés en 2001, le congé de présence parentale (CPP) et l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) sont des dispositifs précieux pour soulager des situations familiales complexes et douloureuses. Ils permettent en effet aux parents d'interrompre leur activité professionnelle tout en bénéficiant d'un revenu afin d'accompagner un enfant dont la dégradation de l'état de santé justifie un accompagnement soutenu. Il peut s'agir d'une pathologie telle qu'un cancer pédiatrique, d'un handicap ou d'un accident particulièrement grave. Pour bénéficier de ces dispositifs, un certificat médical doit attester de la particulière gravité de l'affection et définir la durée prévisible du traitement. Cette durée est censée déterminer celle des droits au CPP et à l'AJPP, dans la limite de trois ans. Force est de constater que les conditions de renouvellement de ces dispositifs sont quelque peu déconnectées de la situation médicale de l'enfant.

la première période de trois ans. Au-delà des cas de rechute ou de récidive, ce renouvellement est de droit en cas de perpétuation de la gravité de l'état de santé. Toutefois, c'est seulement à l'issue de la période initiale de trois ans, et non au sein de cette période, que le renouvellement peut avoir lieu. En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a ouvert la possibilité pour le salarié, avec l'accord de son employeur, de fractionner le CPP ou de le transformer en période d'activité à temps partiel, afin de mieux concilier l'accompagnement de l'enfant et le maintien d'une activité professionnelle. Le recours au CPP et à l'AJPP est dynamique : le nombre de bénéficiaires a augmenté de 70 % sur la période allant de 2013 à 2020. Un peu moins de 10 000 familles en ont ainsi bénéficié en 2020. Alors que le montant de l'AJPP était jusqu'ici revalorisé en fonction de l'inflation,

Je me félicite également du projet de dématérialisation des attestations mensuelles de l'employeur que le bénéficiaire doit produire tous les mois pour renouveler ses droits à l'AJPP. Ce mode de transmission des informations nécessaires aux caisses d'allocations familiales, prévu d'ici à la fin de l'année 2022, devrait faciliter grandement la vie des allocataires. J'en viens au contenu de la proposition de loi déposée par le député Paul Christophe. Son article unique ouvre la possibilité de renouveler le CPP et le crédit d'AJPP au-delà de 310 jours sur la période de référence initiale de trois Cette évolution est pleinement justifiée par le souci de mieux tenir compte de la réalité de la pathologie ou du handicap de l'enfant et des soins qu'il requiert. La possibilité de renouvellement après la période initiale de trois ans, que nous avons votée dans la loi du 8 mars 2019, présente en pratique un En effet, au bout de trois ans, la plupart des enfants sont généralement soit guéris, soit, malheureusement, décédés. Les dispositions actuelles ne répondent donc pas aux besoins des quelque 600 foyers qui, au cours de la période de référence de trois ans, épuisent leur crédit de 310 jours d'AJPP. Dans le cas de cancers pédiatriques, selon les estimations les plus pessimistes, 30 % des parents bénéficiaires de l'AJPP auraient besoin d'une prolongation du nombre de jours d'allocation.

si la santé de leur enfant le requiert. Une amélioration, capitale au titre du principe d'égalité, aurait néanmoins pu être apportée à la proposition de loi. Il semble en effet indispensable d'étendre aux agents publics le bénéfice de ces nouvelles dispositions. Toutefois, cette extension nécessite une modification des lois statutaires des trois fonctions publiques et du code de la défense. Cette extension constituant une dépense supplémentaire, seul un amendement gouvernemental peut y procéder. Pour réparer cet oubli, j'ai exposé à la commission une solution de nature à ne pas compromettre l'adoption rapide de la proposition de loi, dans un contexte d'encombrement de l'ordre du jour parlementaire. Ce texte a en effet été adopté voilà déjà près d'un an par l'Assemblée nationale et nombre de foyers ont épuisé leur crédit de 310 jours et ne peuvent le renouveler.

garantirait aux familles qui arriveraient en fin de droits dans les semaines prochaines la possibilité de renouveler aussi sereinement que possible leur accès au CPP et à l'AJPP.

Mes échanges tant avec le rapporteur de l'Assemblée nationale qu'avec le cabinet du secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles me font penser qu'il s'agit de la solution la plus efficace dans l'intérêt des familles concernées.

afin de permettre au dispositif de mieux répondre aux besoins d'accompagnement de l'enfant. J'identifie, à cet égard, deux enjeux principaux. Le premier enjeu concerne l'équité parentale il nous faut réfléchir aux moyens de garantir aux deux parents la possibilité d'accompagner leur enfant. Le parent dont l'emploi est le plus rémunérateur a en effet tendance à maintenir son activité, laissant l'autre parent, bien souvent la mère, interrompre la sienne afin de se consacrer à l'accompagnement de l'enfant. La situation familiale peut s'en trouver durablement affectée, de la dégradation de l'employabilité du parent accompagnant et du sentiment de culpabilité de l'autre parent n'ayant pu accompagner son enfant autant qu'il l'aurait souhaité. Nous devons ainsi nous interroger sur l'évolution possible des conditions de cumul de l'AJPP entre les deux parents, en les alignant sur celles qui sont aujourd'hui prévues pour l'allocation journalière du proche aidant (AJPA). En effet, deux parents peuvent cumuler, à eux deux, 44 jours d'AJPA par mois. Je forme le voeu qu'il en soit de même à l'avenir pour l'AJPP, dont le bénéfice est aujourd'hui limité à 22 jours par mois pour les deux parents. enjeu concerne la suppression du plafonnement de l'AJPP. Cette question reste ouverte, dès lors que la prise en charge de certaines pathologies, comme les leucémies ou les tumeurs cérébrales, peut justifier un accompagnement parental dépassant les 620 jours. En attendant, il nous faut agir dans l'intérêt immédiat des familles. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'adopter sans modification ce texte, qui répond aux attentes des familles et dont nous devons garantir une entrée en vigueur

le CPP et l'AJPP permettent aux parents d'accompagner un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, lorsqu'ils sont contraints d'interrompre leur activité professionnelle afin d'assurer une présence soutenue auprès de leur enfant. Un salarié peut ainsi bénéficier, au titre du CPP, d'un maximum de 310 jours ouvrés de congé. Ces dispositifs ont été modifiés à deux reprises afin d'en renforcer la flexibilité et de mieux répondre aux besoins d'accompagnement de l'enfant. Ainsi, la loi du 8 mars 2019 a permis d'assouplir les conditions de bénéfice du CPP et de l'AJPP en tenant compte de la durée et des conséquences des traitements. Depuis, ces deux dispositifs permettent d'apporter un soutien aux parents actifs ayant un enfant à charge dont la dégradation de l'état de santé rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. L'AJPP s'élève actuellement à 52 euros pour une personne seule et à 44 euros pour une personne en couple. Cette allocation ne peut être versée que 22 jours par mois, ce qui correspond au nombre de jours ouvrés. Ainsi, un bénéficiaire de l'AJPP reçoit en moyenne 780 euros par mois. L'arrêt de l'activité professionnelle peut donc représenter un sacrifice financier non négligeable, en particulier pour les familles monoparentales. En 2020, un peu moins de 10 000 familles ont bénéficié de l'AJPP, pour un coût total de 97 millions d'euros. Ce nombre est en constante progression- il a augmenté de 6 % en 2019 -, ce qui traduit sans doute une meilleure information des personnes concernées. La possibilité de renouveler les droits au CPP et à l'AJPP est déjà ouverte aux cas de rechute ou de récidive. À l'issue des trois premières années, une nouvelle période de trois ans peut être ouverte, le nombre de jours de CPP et d'AJPP pouvant atteindre un maximum de 310 dans ces deux hypothèses. Par ailleurs, la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité, et non plus pour moitié, dans la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

Actuellement, le CPP et l'AJPP permettent de répondre à la plupart des besoins, puisque le taux de consommation moyen de l'AJPP est de 173 jours, soit un niveau nettement inférieur au plafond en vigueur. Cependant, 6 % des bénéficiaires de l'AJPP, soit environ 600 personnes, utilisent entièrement leurs droits, ce qui laisse à penser que le dispositif n'est pas suffisant pour eux. Il est donc proposé d'apporter une réponse appropriée à ces familles, qui ont besoin de plus de 310 jours sur les trois premières années. des professionnels et le droit à l'oubli de Mme Nathalie Elimas, il était déjà prévu d'apporter une réponse à ce problème en supprimant le plafond de 310 jours en cas de cancer pédiatrique. Malheureusement, l'amendement gouvernemental adopté lors de la discussion à l'Assemblée nationale a simplement permis d'étendre les possibilités de réouverture des droits au CPP et à l'AJPP à l'issue de la période initiale des trois ans, non pas d'allonger la durée des droits au cours de la période initiale de trois ans. Aussi le droit actuel n'est-il pas pleinement satisfaisant, car il existe des situations nécessitant un accompagnement long et continu de l'enfant au-delà de 310 jours au cours des trois premières années de la maladie, comme dans le cas des cancers pédiatriques. L'article unique de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à ces situations. Il prévoit la possibilité de renouveler une fois la durée maximale du CPP et de l'AJPP avant la fin de la troisième année suivant l'ouverture des droits. Ce renouvellement sera possible avant la fin du terme initialement fixé et conditionné à la délivrance d'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant,

pourra bénéficier de manière continue de deux fois plus de jours pour poursuivre l'accompagnement de son enfant, soit un total de 620 jours. Le coût de ce dispositif devrait s'élever à 6,2 millions d'euros par an. Il permettra de faire passer de quatorze à vingt-huit mois la durée continue maximale du CPP et de l'AJPP à temps plein. Un parent pourra ainsi bénéficier en continu de 620 jours de CPP et d'AJPP. Ces nouveaux droits pourront être consommés au cours d'une nouvelle période de trois ans. Le groupe Les Républicains est favorable à cette mesure, qui renforce le soutien aux familles qui traversent une épreuve si difficile. Il soutiendra ce texte, dont je salue l'initiative.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires accueille favorablement ce texte, qui permettra de mieux répondre aux besoins des familles confrontées à des situations exigeant un accompagnement soutenu d'un enfant malade et ayant épuisé les droits aux allocations journalières et aux jours de congés afférents.

Elle a pour objectif de mieux couvrir les besoins non satisfaits de parents en souffrance, auxquels on a quelquefois tenté de répondre par la solidarité entre salariés, ce qui ne pouvait raisonnablement se substituer à une majoration du dispositif. été rappelé, les parents peuvent bénéficier au maximum de 310 jours de congé de présence parentale et d'allocations journalières de présence parentale, dans la limite d'une durée de trois Le texte permet de renouveler le versement de l'allocation durant un maximum de 310 jours au cours d'une nouvelle période de trois ans, sans attendre la fin du terme de la première période de trois

nous tenons à soulever quelques points qui méritent vigilance. Tout d'abord, les parents ne doivent pas être contraints de recourir à la prolongation du dispositif faute de réponses institutionnelles de qualité.

c'est le parent dont l'emploi est le plus rémunérateur qui se maintient en général en activité, laissant l'autre parent- bien souvent la mère -interrompre son activité afin de se consacrer à l'accompagnement de l'enfant

Cette loi fait avancer la société, mais nous devons parallèlement rendre effective l'égalité salariale, si nous voulons dépasser l'impuissance devant le constat d'un congé pris uniquement par les mères, renforçant la persistance de rôles parentaux différenciés. La parole

Si le congé de présence parentale et l'allocation journalière de présence parentale permettent de soulager des situations familiales complexes et douloureuses, ces dispositifs comportent des limites. Actuellement, les quelque 600 foyers qui épuiseront bientôt leur crédit de 310 jours d'indemnisation perdront le droit à l'allocation journalière de présence parentale. Cette proposition de loi apporte donc une réponse en ouvrant la possibilité de renouveler le congé de présence parentale et l'allocation journalière correspondante au-delà des 310 jours sur une période de trois Cette mesure est positive, car elle permet de mieux tenir compte de la réalité de la pathologie ou du handicap de l'enfant et des soins qu'il requiert. Nous aurons peut-être l'occasion d'aller plus loin lors de l'examen, au mois de décembre en créant un congé spécifique. La proposition de loi que nous discutons aujourd'hui m'offre la possibilité d'évoquer le montant insuffisant de l'indemnisation journalière. Nous nous félicitons de la revalorisation au niveau du SMIC du montant de l'allocation journalière du proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale. Toutefois, plus globalement- nous aurons l'occasion d'en discuter lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 la semaine prochaine -, nous militons pour le rétablissement des cotisations patronales à la branche famille, pour garantir une indemnisation à 100 % des congés parentaux. Au-delà du niveau de l'indemnisation des congés parentaux, ce sont les conséquences de la suspension du contrat de travail qui posent problème à de nombreuses personnes qui nous interpellent dans nos territoires, comme l'a souligné Cathy Apourceau-Poly en commission. Actuellement, lorsqu'un salarié décide de prendre un congé de proche aidant, il perd non seulement son salaire, mais également le bénéfice des cotisations associées, ce qui signifie une perte de droit pour sa retraite future. Il n'est pas inutile ici de rappeler qu'il s'agit en majorité Pour pallier cet inconvénient, la loi prévoit une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. Cette affiliation n'étant toutefois pas automatique, nombreux sont ceux qui n'entreprennent pas les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales et qui perdent ainsi leurs droits à la retraite future, ce qui est une forme de double peine. Je tiens, monsieur le secrétaire d'État, à appeler votre attention sur ce sujet, afin que le Gouvernement puisse s'en saisir. En outre, il me semble que cette proposition de loi concernant les enfants et les cancers pédiatriques fait écho à l'actualité de la saturation des urgences pédiatriques. Je pense par exemple aux urgences pédiatriques de Douai, qui avaient annoncé leur fermeture partielle les jours fériés, les week-ends et les soirs de semaine, en raison du manque de pédiatres pour assurer les gardes. Depuis le 15 septembre dernier, ces urgences ont réussi à rouvrir le soir, mais seulement jusqu'à 21 heures. Comment améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant qui souffre d'une pathologie nécessitant un accompagnement, mais qui ne bénéficie pas d'un accès aux soins suffisant ? le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, mais c'est parce que le système craque et que nos réponses ne peuvent pas être partielles qu'il est nécessaire de mettre un oeuvre un plan pluriannuel d'investissement massif dans la santé, qui repose sur des recrutements et une revalorisation salariale, pour rendre ces filières attractives. Il faut également poursuivre les efforts en matière de recherche contre ces cancers. En ce sens, l'amendement de 20 millions d'euros, adopté à l'Assemblée nationale dans

je tiens à remercier le groupe Les Indépendants - République et Territoires d'avoir inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour de nos travaux et je salue la clarté du rapport remis par Colette Mélot.

Les débats dans notre société autour de la place des proches aidants, du temps qu'ils peuvent consacrer aux plus vulnérables et du soutien que l'État peut leur apporter sont de plus en plus prégnants. Cela commence d'abord par la reconnaissance des besoins, puis par la mise en place de dispositifs adaptés, notamment financiers. Modifier le droit en vigueur pour augmenter le nombre maximum de jours de congé de présence parentale adapter les conditions d'octroi de l'allocation journalière de présence parentale sont des mesures pragmatiques pour permettre aux parents d'accompagner de manière soutenue leur enfant, frappé par la maladie ou un accident grave et nécessitant un accompagnement soutenu. soutenu. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui témoigne d'une avancée significative, qui s'inscrit dans la lignée l'une histoire récente.

du 8 mars 2019 a simplifié la vie des parents, en permettant la prise en charge des cancers pédiatriques et le réexamen de la durée prévisible de traitement de l'enfant.

La disposition prévue par cette proposition de loi est parfaitement justifiée et s'applique dans le cas où la santé de l'enfant le requiert et que le bilan médical l'approuve.

En revanche, même si nous voterons ces dispositions afin qu'elles puissent entrer en vigueur dans les plus brefs délais, nous regrettons, comme l'a souligné notre rapporteure, plusieurs limites du dispositif transmis par l'Assemblée nationale.

Mes chers collègues, la détresse des parents face à un enfant touché par la maladie, la pathologie, le handicap ou un accident particulièrement grave ne devrait pas faire de distinction entre le secteur public et le secteur privé.

dans la mesure où elle tend à permettre à la puissance publique d'ajuster des dispositifs qui améliorent les conditions d'accompagnement de familles dans des situations de détresse tout à fait particulières. Pour mémoire, les dispositifs en question, le congé de présence parentale et l'allocation journalière de présence parentale, constituent un soutien pertinent aux actifs ayant un enfant dont l'état de santé implique une présence soutenue

Dans le cas où la gravité de la pathologie de l'enfant nécessite un allongement de ces dispositifs, les parents ont la possibilité de renouveler leurs droits à l'issue de ces trois années, sous réserve de l'accord des équipes médicales concernées. En l'état actuel de la situation, 10 000 personnes bénéficient de ces dispositifs, avec un taux de consommation moyen de 173 jours. Je rappelle néanmoins que 6 % d'entre eux utilisent entièrement leurs droits, ce qui laisse supposer au législateur que ces dispositifs ne seraient pas suffisants pour eux. Ce texte leur apporte une réponse appropriée en permettant, par dérogation au dispositif actuel, d'enclencher le renouvellement de leurs droits avant l'expiration du délai de trois ans.

d'État, j'appelle votre attention sur l'importance de bien, ou de mieux informer les familles de l'existence des dispositifs que nous examinons aujourd'hui. Il serait intéressant de systématiser la redirection des familles par les assistantes sociales, le corps médical ou les psychologues vers des sources telles que le site www.monenfant.fr, qui rassemble de nombreuses informations claires et utiles aux parents.

un souci évident d'égalité et d'efficacité à l'égard de nos concitoyens. Quoi qu'il en soit, notre groupe soutient pleinement cette proposition de loi qui est nécessaire et, naturellement, la votera à l'unanimité.

Ces dispositifs sont en effet essentiels pour permettre aux parents d'interrompre leur activité professionnelle lorsque leur enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un grave accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. bénéficie ainsi à quelque 10 000 personnes chaque année et l'allocation journalière de présence parentale, qui s'élève actuellement à 52 euros pour une personne seule et à 44 euros pour une personne en couple, est versée 22 jours ouvrés par mois. Cette allocation, bien qu'elle soit précieuse pour les familles, ne suffit évidemment pas à compenser la perte financière que représente l'arrêt ou la diminution de l'activité professionnelle de l'un des parents.

aller plus loin, mais cela constitue déjà une revalorisation souhaitable, en particulier en direction des familles monoparentales. La loi du 8 mars 2019 visant à renforcer

Les cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant ont également été pris en compte et la loi a instauré une obligation d'information des organismes débiteurs des prestations familiales quant aux critères et conditions d'attribution de l'allocation journalière aux modalités de demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, dont la prestation de base est cumulable avec l'allocation journalière de présence parentale, et de la prestation de compensation du handicap. La durée du congé de présence parentale est en outre désormais prise en compte en totalité, et non plus pour moitié, dans la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le recours à ce dispositif pourrait par ailleurs s'accroître du fait de la possibilité instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 de fractionner le congé de présence parentale et de le rendre compatible avec une activité professionnelle à temps partiel. Face à la dégradation de l'état de santé d'un enfant, qui conduit bien souvent l'un des parents à arrêter totalement son activité professionnelle, cette mesure permettra de favoriser, autant que possible, le maintien de cette activité et ainsi de préserver le niveau de vie des foyers concernés, déjà durement éprouvés. Ces mesures semblent aujourd'hui satisfaire la majorité des situations individuelles, puisque le taux de recours moyen à l'allocation journalière de présence parentale est de 173 jours, soit un niveau inférieur au plafond de 310 jours en vigueur. vigueur. Une carence du dispositif a cependant été mise en exergue concernant les 6 % des bénéficiaires qui utilisent entièrement ces 310 jours et qui doivent attendre l'expiration d'un délai avant de pouvoir prétendre à leur renouvellement. Cette contrainte temporelle n'est pas en phase avec la réalité vécue par des parents confrontés à une longue pathologie de leur enfant et dont le besoin d'accompagnement est requis de manière immédiate et continue.

sous réserve de la transmission d'un nouveau certificat établi par le médecin qui suit l'enfant et d'un accord explicite du service du contrôle médical. Un parent ayant épuisé les 310 jours octroyés pourra donc bénéficier sans délai d'un nouveau contingent de 310 jours, afin de poursuivre l'accompagnement de son enfant.

Si nous partageons le souhait d'une adoption conforme de ce texte en vue d'une mise en oeuvre rapide en direction des familles concernées, je souhaite néanmoins insister sur la nécessité de respecter, dans le même temps, les engagements pris sur plusieurs sujets : d'abord, la réduction des délais d'instruction des dossiers et la dématérialisation de la transmission aux caisses d'allocations familiales des informations nécessaires au versement de l'allocation journalière

l'importance de renforcer l'information des familles quant à l'existence de ces dispositifs qui restent encore trop souvent méconnus, même si le recours au congé de présence parentale et à l'AJPP tend aujourd'hui, fort heureusement, à s'améliorer. Nous renouvelons donc notre plein soutien à ce texte qui est accueilli très favorablement par les familles, les aidants et les associations qui leur viennent en aide dans ce combat au long cours. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, améliorer la situation des familles dont les enfants sont atteints de cancer et celle des familles dont les enfants souffrent d'autres pathologies nécessitant des soins lourds et de très longue durée, tel est l'objectif de la proposition de loi que notre assemblée examine aujourd'hui. Adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale il y a presqu'un an jour pour jour, ce texte traite d'une problématique qui est au coeur du quotidien de milliers de familles. Je salue la présence dans nos tribunes du député Paul Christophe,

Nous sommes nombreux à avoir en mémoire un ami, un membre de notre famille ou un collègue de travail touché par cette situation. En tant que parents, nous ne pouvons qu'imaginer leur souffrance, leur dévouement, leur ténacité pour soutenir et accompagner leur enfant. Il appartient donc au législateur de permettre une présence renforcée des parents auprès de leur enfant atteint d'une pathologie et de faire en sorte que cette situation, déjà d'une extrême difficulté, puisse être surmontée dans les meilleures conditions possible.

Ce droit à 310 jours peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie de l'enfant, seulement une fois que la période de trois ans est écoulée. Or, dans certains cas- je pense tout particulièrement aux enfants atteints d'un cancer -, le droit actuel ne semble pas suffisamment adapté à la présence et à l'accompagnement nécessaires dans le cadre Comment expliquer à un parent dont l'enfant est toujours malade qu'il doit attendre plusieurs mois avant de pouvoir obtenir de nouveaux jours et de nouveaux droits ? Partant de ce constat et guidés par la volonté de sécuriser la situation des familles, proposition de loi entendent ouvrir la possibilité, sous certaines conditions, de renouveler le versement de l'allocation pour une durée maximum de 310 jours et pour trois ans supplémentaires, sans attendre le terme de la première période de trois ans. Nous partageons pleinement cet objectif. Les maladies telles que le cancer ou d'autres pathologies nécessitant des soins lourds et de très longue durée demandent un accompagnement soutenu, essentiel pour surmonter la maladie de l'enfant. Les difficultés qu'une famille rencontre face à la maladie ne doivent pas être aggravées par des problèmes financiers. Le soutien à ceux qui en ont le plus besoin est au coeur de nos valeurs de solidarité et de fraternité. Cette double peine induite par le dispositif en vigueur se devait d'être corrigée.

Je salue ensuite le travail réalisé par le passé, qui a déjà permis de répondre en grande partie aux besoins des patients et de leurs parents. Je citerai ainsi la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux,

À l'âge de 9 ans, cet enfant a déclaré une maladie orpheline qui se révélera mortelle. Le père était agriculteur, la mère enseignante. Pour accompagner son enfant dans les derniers moments de sa vie, la mère a fait une demande de quelques jours de disponibilité à l'éducation nationale : ce n'était pas dans les usages et cette demande lui a été refusée. Les règles étaient alors trop rigides et aucun dispositif de congé n'existait à l'époque pour permettre à un père ou à une mère de quitter son travail quelques jours, voire quelques semaines, pour rester auprès d'un enfant gravement malade. Cette tragédie familiale et bien d'autres situations similaires montrent l'importance de la proposition de loi déposée par le député du Nord Paul Christophe. texte est le fruit d'une expérience personnelle et d'un parcours politique marqué par un engagement continu, dans le dessein de bâtir une société plus juste, plus humaine et plus solidaire.

Cette proposition de loi améliore le dispositif de congé pour présence parentale, en permettant au salarié dont l'enfant est atteint d'une grave maladie de se rendre disponible pour l'accompagner. Ce congé est associé à une allocation journalière versée au maximum 310 fois sur une période de trois ans, allocation qui verra son montant revalorisé au niveau du SMIC dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, tout comme le montant de l'allocation journalière du proche aidant. La question de la suppression du plafonnement a été évoquée lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, Le gouvernement avait alors proposé d'assouplir les conditions de renouvellement de ce congé, dans deux cas de figure- après trois ans ou avant trois ans -, à condition que le plafond des 310 jours de congé n'ait pas été atteint. sécurité sociale pour 2020 a autorisé l'utilisation fractionnée de ces congés, contribuant à une meilleure souplesse du dispositif. Cependant, le congé de présence parentale reste imparfait pour une partie des bénéficiaires, lorsque la maladie de l'enfant nécessite une présence soutenue de l'un de ses parents plus de 310 jours en trois ans. En effet, le renouvellement de ce congé est actuellement impossible lorsque l'ensemble des jours de congé a été consommé sur cette période. Cette situation concerne environ 6 % des bénéficiaires, soit 600 familles chaque année. La proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu s'adresse à ces familles, lesquelles sont parmi les plus vulnérables.

d'un handicap ou d'un accident grave. Leur enfant ayant besoin d'une présence soutenue et de soins contraignants, ces parents n'ont parfois pas d'autre choix que d'interrompre leur activité professionnelle. Il est alors indispensable que la solidarité nationale vienne compenser la perte de revenus qui en découle. La question centrale qui les préoccupe est celle de la durée du congé et du versement de l'allocation : elle est actuellement de 310 jours sur une période de trois ans après le début de la maladie, ce qui reste insuffisant. Bien que la loi du 8 mars 2019 ait permis de renouveler les droits du congé et de l'allocation au-delà de trois ans, le dispositif en vigueur n'est toujours pas en phase avec les réalités que connaissent certaines familles. Prenons le cas des 2 500 cas de cancers pédiatriques dénombrés chaque année. Après deux ou trois années de traitement, l'enfant est souvent soit guéri, soit malheureusement décédé- cela représente 20 % des cas -, ce qui rend sans effet la possibilité existante de renouvellement. La possibilité de réouverture des droits en cas de rechute ou de récidive de l'enfant n'est pas toujours garantie aux familles, qui se heurtent parfois au refus des CAF, le versement de la prestation étant soumis à l'avis favorable du service du contrôle médical. Les formalités sont également trop lourdes, la prestation étant, de l'avis même de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), complexe à mettre en oeuvre. Devant la détresse de ces familles, nous ne pouvons que saluer et soutenir la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, car elle vise à leur permettre de renouveler une fois la durée maximale du congé et de l'allocation avant la fin de la période de trois ans, et non plus seulement au terme de celle-ci. Par cette mesure de justice sociale, le législateur prend mieux en compte la réalité de la pathologie ou du handicap de l'enfant et des soins qu'il requiert.

et son extension aux conjoints collaborateurs d'une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole. Un bémol toutefois : l'éparpillement de ces mesures portant sur un même sujet dans des textes différents nuit considérablement à la lisibilité de la réforme. Regrettons également que le nouveau dispositif de la proposition de loi ne s'applique pas aux agents publics, alors même que chacune des lois relatives aux trois fonctions publiques prévoit le bénéfice du congé parental et aurait donc également mérité d'être modifiée en ce sens.

qui décide d'interrompre son activité afin de se consacrer à son enfant. Cette situation contribue à dégrader l'employabilité du parent accompagnant et à aggraver le sentiment de culpabilité de l'autre parent, qui ne peut pas participer à l'accompagnement autant qu'il l'aurait souhaité. Or un enfant malade a besoin du soutien quotidien de ses deux parents. Mes chers collègues, nous discutons d'un sujet complexe et douloureux pour les familles. Je ne peux m'empêcher de souligner le manque d'attention dont sont parfois victimes les parents d'enfants malades dans leur environnement professionnel. Permettez-moi de citer l'exemple vécu par l'une de mes proches, interne en médecine, qui s'est vu refuser un transfert de stage dans l'hôpital où était soigné son bébé de deux mois, atteint d'un cancer, au motif que cela créerait un précédent et pourrait entraîner des demandes multiples d'autres internes ... Espérons qu'il n'y ait pas de nombreux internes ayant des enfants atteints de cancer ! Ce genre de réponse n'est pas acceptable. La situation de l'enfant doit primer sur toute autre considération. La bienveillance doit l'emporter sur l'indifférence. Malgré les imperfections qu'il contient, la commission des affaires sociales a voté le texte sans modification afin de répondre aux situations d'urgence de certains foyers fragilisés par la crise sanitaire. nombreuses familles ayant déjà épuisé leur crédit de 310 jours, il est en effet indispensable d'adopter rapidement ce nouveau dispositif, un vote conforme du Sénat, même si ce vote ne doit pas exonérer le Gouvernement d'intervenir dans les meilleurs délais pour en corriger les failles. Le groupe Les Républicains votera donc en faveur de cette proposition de loi. La parole est

la proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Mes chers

est suspendue. La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée l'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, ont été publiées.

pays, particulièrement en France, où la Nation s'est construite grâce à l'État. L'administration d'un pays fait partie de son identité. Toute tentative visant à moderniser l'administration laisse un goût d'inachevé, d'abord parce que l'administration vit avec son temps et en partage autant les nouveautés que les archaïsmes, ensuite, parce que l'administration est à l'image du pays et en partage autant les qualités que les défauts. En revanche, il est sain que le législateur cherche toujours à rendre son fonctionnement aussi intelligible que possible, du point de vue des administrés et non de celui des administrateurs.

réside à mes yeux tout l'intérêt du principe selon lequel « silence gardé par l'administration vaut acceptation », qui constitue un moyen simple et efficace de s'assurer que la puissance publique réponde effectivement aux attentes des citoyens.

dès le début, il y avait deux fois plus de procédures administratives dérogatoires que de procédures relevant du principe général. En d'autres termes, dès le début, l'exception était la norme et le principe général de la loi était largement dévoyé.

Ces exceptions laissent les coudées franches au Gouvernement pour déroger au « silence vaut acceptation », ce qui nuit à la force de ce principe établi par le législateur. Il s'agit précisément du sujet dont nous allons débattre aujourd'hui. je vous propose de redonner sa vigueur au principe général, en limitant la possibilité d'y déroger par voie réglementaire et en harmonisant les délais dérogatoires. L'idée est de rendre le système plus lisible pour les usagers. Le dispositif de la proposition de loi se fonde sur un constat réalisé sur le terrain auprès des acteurs qui entreprennent et sont à l'initiative- bref, de tous ceux qui veulent faire changer les choses.

J'insiste : je ne fais ni mauvais procès ni mauvaises généralisations. Nous connaissons tous des serviteurs de l'État qui exercent avec beaucoup de professionnalisme et qui font preuve d'une grande réactivité. Ils font honneur à la fonction publique, et je tiens à les remercier. ! Je tiens tout de même à vous raconter une anecdote qui en dit long sur les effets néfastes du « silence vaut rejet ». Dans mon territoire, un entrepreneur engage une démarche auprès d'une administration pour réaliser un projet. Plusieurs mois passent et cette demande demeure sans réponse. L'entreprise relance l'administration. Là encore, pendant plusieurs mois, l'administration reste aux abonnés absents. Une troisième tentative vaine. La situation dure pendant deux ans. L'entrepreneur choisit donc d'engager son projet et de prendre les devants pour faire bouger les choses. Là, ni une ni deux, l'administration se réveille et sanctionne l'entreprise. Malheureusement, un tel scénario n'a rien d'exceptionnel. Si les entrepreneurs bloqués par l'administration ne représentent qu'une minorité des usagers, ils demeurent trop nombreux pour que nous ne fassions rien. Bien évidemment, la situation est encore pire pour les usagers qui se retrouvent démunis face à la complexité administrative et qui ne disposent d'aucune aide juridique pour s'y retrouver. Nous devons leur simplifier la vie. Au cours de ce quinquennat, plusieurs textes ont été défendus par le Gouvernement et votés par le Sénat, afin de simplifier les relations entre les citoyens et l'administration. Je pense notamment à la loi de 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Essoc).

L'article 72 de la loi Essoc prévoyait que le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement pour faire le point sur l'application du principe « silence vaut acceptation ». Dans ce rapport, le constat demeure sans appel seulement un tiers des procédures administratives respecte le principe général. En d'autres termes, l'exception demeure la norme et le pouvoir législatif n'a plus la main pour faire appliquer le principe général. la loi Essoc a été une occasion manquée d'adopter des propositions concrètes et nous avons dû nous contenter d'un rapport remis par le Gouvernement. Ce rapport indique également

Je tiens à alerter l'opinion sur ce point, car tout porte à croire que la situation en la matière risque de se détériorer dans les prochaines années. La prise en compte des enjeux écologiques ne doit pas entraver les initiatives individuelles. Je crois sincèrement que nous devons fonder la relation entre les usagers et l'administration sur la confiance mutuelle plutôt que sur la défiance réciproque. Le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP),

Les propositions qu'elle défend au nom de la commission des lois vont dans le sens de notre texte, et je m'en réjouis. Je suis heureux que nous en débattions avec l'ensemble des groupes de façon constructive, pour trouver une solution de consensus.

Depuis lors, le silence de l'administration vaut en principe acceptation, sous réserve de très nombreuses exceptions prévues par le droit. Si l'objectif de cette réforme de multiplier les procédures de SVA a été rempli - elles ont été multipliées par quatre force est de constater que ce résultat a été obtenu en sacrifiant la lisibilité du régime du silence de l'administration prévu par le code des relations entre le public et l'administration. En effet, l'inversion du principe s'est accompagnée de la création d'une multitude d'exceptions qui rendent la compréhension du droit positif assez chaotique. la ferme des mille vaches en est une preuve, puisqu'il a fallu un pourvoi en cassation et une décision du Conseil d'État pour déterminer si, en l'espèce, le silence de l'administration valait acceptation ou rejet. Autre preuve, même l'administration en charge de la publication de la liste des procédures de SVA a du mal à s'y retrouver ... Alors, mettez-vous à la place de l'usager lambda

Si vous demandez à une administration d'effectuer un choix parmi plusieurs possibilités, son silence ne permettra pas de répondre à la question De la même manière, si vous demandez à une administration de vous verser une indemnité, son silence n'entraînera pas le versement de la somme demandée.

la perte d'un courrier ou une erreur de traitement aboutit à l'acceptation tacite d'une demande par l'administration, même si l'usager ne remplit pas les critères d'attribution. se retrouve donc dans une situation plus favorable qu'une personne présentant le même dossier et ayant été déboutée à juste titre. Il y a donc un problème de

De trop nombreuses divergences nous ont conduits à ne pas adopter de texte en commission, en application du d'usage pour les propositions de loi de niche.

Les relations entre le public et l'administration sont perçues comme des relations purement bilatérales, souvent conflictuelles. conflictuelles. Or l'activité de régulation confiée aux administrations a pour objet de préserver l'ordre public, l'environnement et les droits des tiers. L'instruction d'une autorisation d'urbanisme peut, par exemple, révéler une atteinte possible à une servitude établie au bénéfice d'un tiers. L'administration n'est pas l'ennemie de l'usager, il est important de le rappeler. Tout à fait ! Partant de ce constat, notre second principe directeur réside dans le maintien d'un équilibre entre les conditions d'une bonne administration et les droits du public.

SVA, nous avons préféré conserver cette faculté tout en précisant les cas dans lesquels une telle dérogation demeurait possible. En revanche, nous émettrons un avis favorable sur l'amendement déposé par Jean-Pierre Sueur qui a pour objet de réécrire l'article 4 afin de plafonner les délais dérogatoires fixés par le pouvoir réglementaire pour établir les décisions implicites de l'administration. Ce plafonnement semble nécessaire pour sauvegarder l'intérêt des usagers et éviter que des délais exagérés ne vident de son sens le principe SVA. La recherche d'équité dans les rapports entre l'administration et le public a également orienté la réécriture de l'article 5 que nous vous proposerons. prévoit que les appels de pièces complémentaires suspendront simplement les délais laissés à l'administration pour instruire les demandes, ne permettant plus de remettre les compteurs à zéro. En effet, certaines administrations détournent les demandes de pièces complémentaires, dans le cadre d'une manoeuvre dilatoire visant à allonger significativement le délai dont elles disposent avant qu'une décision implicite d'acceptation soit rendue. Outre ces trois modifications importantes, nous vous proposerons la suppression totale ou partielle d'articles présentant certaines malfaçons et pour lesquels des modifications ne nous ont pas semblé possibles ni souhaitables. l'adoption de ces différents amendements, nous vous engageons à adopter cette proposition de loi. Ainsi modifiée, elle nous semble constituer la garantie d'un meilleur équilibre entre les intérêts de l'administration et ceux de l'usager. La parole est

mesdames, messieurs les sénateurs, le Président de la République a fixé à chacun de ses ministres un objectif très clair : garantir la culture de la bienveillance et de l'efficacité dans l'administration au service des usagers, simplifier les démarches administratives, réduire les délais de réponse aux administrés et instaurer une relation de confiance entre les citoyens et leurs services publics. C'est aussi ma feuille de route, en tant que ministre de la transformation et de la fonction publiques.

sur ce sujet essentiel. Je me réjouis que nous ayons ce débat aujourd'hui pour aborder un point de la vie quotidienne de nos concitoyens : la nature de leurs relations avec l'administration. Dans votre exposé des motifs, vous appelez de vos voeux des relations entre les citoyens et la puissance publique fondées sur la confiance et le dialogue. Vous insistez sur l'importance d'une inversion de la logique de l'action publique, en partant des besoins du citoyen et non de ceux de l'administration. Ces objectifs, le Gouvernement les partage pleinement. Depuis la création de mon ministère, j'ai souhaité que les administrations et leurs agents soient davantage tournés vers les usagers et arrêtent de piloter leur action en vase clos.

Nous ne pouvons pas nous résoudre aux inégalités existant, dans l'accès aux droits, entre nos concitoyens et qui résultent de ces complications. Cela passe d'abord par la restauration d'un lien de confiance entre l'usager et l'administration, une confiance

depuis 2018, près de 335 000 droits à l'erreur ont été accordés à des usagers et 2 millions d'erreurs administratives détectées de manière proactive par l'administration n'ont pas conduit à des pénalités, mais ont été simplement résorbées, clarifiées. si des erreurs de bonne foi peuvent intervenir, c'est bien souvent parce que notre réglementation et nos procédures sont complexes. Si le droit à l'erreur en atténue les effets, la simplification- autre bataille que je mène -en traite les causes.

inférieur à quinze jours. Nous travaillons également à la numérisation complète de la procédure de dépôt et de traitement des demandes de permis de construire et d'autorisations d'urbanisme dans les communes de plus de 3 500 habitants

qui permet à chaque usager de partager son expérience dans ses relations avec l'administration, de donner son avis, donc de guider l'amélioration du service public. En un an, nous avons reçu 3 millions d'avis d'usagers et 3 000 personnes ont pris le temps de raconter précisément leur expérience et de proposer des améliorations concrètes de démarches administratives ou de souligner la qualité d'un service et des liens tissés avec l'administration.

en lien avec les agents publics, qui sont les premiers acteurs de cette action, que nous cherchons à rendre plus efficace et plus proche des Français. Nous avons encore beaucoup à faire en la matière et je sais que nous pourrons travailler ensemble à l'amélioration du quotidien de nos concitoyens, mais, à l'heure où tous nous disent, souvent avec raison,

Ce concept, quoique récent, est familier à tous. Il s'est imposé au fur et à mesure comme une solution d'équilibre entre l'administration et les usagers, comme une simplification nécessaire et bienvenue. encadré depuis 2013, passé un certain délai, une absence de réponse de la part de l'administration doit être considérée comme un accord. Toutefois, ce principe reste très limité dans sa mise en oeuvre et, comme notre rapporteur a pu le rappeler, il ne présente pas que des avantages. L'un des inconvénients intrinsèques mis en avant est celui de la publication des décisions, permettant notamment d'ouvrir droit à des recours par des personnes tierces. En effet, la publicité dans l'action de l'administration, comme d'ailleurs dans notre action de législateur, qui contribue à ce que certains appellent désormais la transparence, est essentielle. L'équilibre nouveau recherché entre l'administration et l'administré ne saurait se faire aux dépens de l'équilibre général et de l'ordre public ni mener à la privation de droits de certains. Une autre faiblesse réside aussi évidemment dans les inévitables problèmes matériels des demandes, comme un courrier perdu. Une Une difficulté majeure engendrée par la mise en oeuvre de ce principe est finalement relative à sa lisibilité : délais variant d'une administration à l'autre, nombreuses exceptions possibles ou encore interprétation variable des tribunaux lors d'un recours sur l'applicabilité ou non de ce principe. Sur ce dernier point, les travaux de qualité de notre rapporteur ont mis en relief les difficultés liées à « la distinction entre acte réglementaire et décision individuelle[, qui] n'est pas toujours parfaitement claire pour certains actes Toutefois, ce principe oblige l'administration ; il l'oblige à instruire ou non des demandes légitimes des citoyens et il crée une sorte de sanction en cas de manquement dans cette instruction. Il permet aussi de ne pas pénaliser l'usager, que celui-ci soit une personne privée ou une entreprise, pour les retards de l'administration, lorsque son action dépend de cette décision. Clairement, cette proposition de loi est motivée par une ambition sérieuse et louable de simplification et d'efficacité dans les relations entre usagers et administration, mais la rédaction parfois trop large de certains articles nous appelle à quelque prudence. Vous connaissez l'attention que nous portons au pouvoir local des maires, comme nous l'avons défendu lors de l'examen nous sommes bien conscients de leur besoin d'accompagnement, d'ingénierie ou de conseil dans certains domaines. Il reste important de développer l'aide et l'appui technique de l'administration centrale et des services déconcentrés auprès des plus petites communes, afin que celles-ci puissent faire face aux demandes nombreuses et variées.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nul n'est censé ignorer la loi. Cet adage simple cache une réalité complexe, puisque les citoyens sont en permanence

par exemple, les précisions et détails qui devraient être inscrits dans la loi pour traduire l'ensemble des dérogations. C'est pourquoi nous défendons, à l'instar de nos collègues, une solution d'équilibre

Cela étant, nous ne pouvons appréhender la complexification des rapports entre l'administration et les citoyens au travers de cette seule approche, sans en évoquer les raisons structurantes. Depuis plusieurs mandats présidentiels, les administrés subissent des privatisations, mutualisations et fermetures de services publics.

En déléguant les services publics, les différents gouvernements ont mis ces derniers au service du profit et non plus de l'intérêt général., la proximité et le temps sont des gages d'efficacité, qui impliquent inévitablement des moyens humains et financiers. Investir dans les services publics en rendant ceux-ci plus accessibles

cette proposition de loi vise à renforcer le principe législatif selon lequel le silence gardé par l'administration vaut acceptation. Ce principe général, établi par la loi du 12 novembre 2013, s'applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l'État et de ses établissements publics depuis le 12 novembre 2015, aux demandes adressées aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d'un service public administratif. Le constat est simple : le principe général posé par la loi est affaibli par de très nombreuses exceptions d'origine réglementaire. Le rapport remis le 1 avril 2019 par le Gouvernement au Parlement en témoigne : « si l'on prend en compte l'ensemble des procédures recensées par les ministères, le taux

est d'améliorer la réactivité des services administratifs. Nous ne pouvons que cautionner cette démarche : la confiance doit être la pierre angulaire des relations entre l'administration et les administrés.

La nouvelle rédaction de l'article 1, proposée par voie d'amendement par Mme le rapporteur, encadre plus étroitement les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut exclure l'application du silence vaut acceptation. Cette rédaction de compromis nous semble excellente. À l'article 2, qui prévoit la publication de deux listes distinctes,

Le silence ne saurait donc constituer l'expression d'une volonté positive, de sorte que l'inertie de l'administration révélait alors l'absence de décision et le refus d'exercer la fonction. Un peu plus d'un demi-siècle plus tard, dans une décision du 26 juin 1969, le jeune Conseil constitutionnel énonçait encore « que d'après un principe général de notre droit le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet et, qu'en l'espèce, il ne peut y être dérogé que par une décision législative Cette mise en perspective nous dit bien le bouleversement qu'a représenté la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, qui a marqué une rupture symbolique : le silence de l'administration devrait désormais valoir acceptation.

qu'en réalité il n'y avait plus, s'agissant du sens du silence de l'administration, ni principe ni exception. Chaque procédure administrative est dans une catégorie particulière.

Avec quelques années de recul, il faut admettre que ce nouveau régime peine toujours à être satisfaisant. Il a trop perdu de vue l'esprit de simplification qui était le sien dans les rapports entre administration et usagers.

Bien sûr, chercher à résoudre les difficultés que pose l'application du principe « silence vaut acceptation » est une tâche ardue- cela a été souligné lors de l'examen du texte en commission.

Madame la ministre, dans le cadre de la réhumanisation de vos rapports avec nous, quelles conséquences allez-vous en tirer ? Sur ces deux textes, allez-vous saisir l'Assemblée nationale pour que le débat se poursuive ou allez-vous

! Je sais bien que le « en même temps » est à la mode, mais on ne peut conjuguer la verticalité perpétuelle avec la réhumanisation dont vous parlez. La parole

Les objectifs de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui sont honorables et personne, à la lecture de l'exposé des motifs, ne pourrait s'inscrire en sa défaveur. Cependant, il existe un écart entre cet exposé et la réalité technique du dispositif législatif prévu.

lisibilité du droit pour les usagers. Les faiblesses intrinsèques à ce principe n'ont jamais été surmontées et posent aujourd'hui difficulté. Comme l'a souligné Mme le rapporteur, que je salue pour la qualité du travail réalisé, les sept articles proposés par notre collègue posent quelques difficultés d'ordre technique. Ainsi, l'existence de deux listes distinctes prévue à l'article 2 pourrait pénaliser certaines administrations, notamment celles des collectivités territoriales, alors même qu'elles n'ont pas la charge de leur publication, ce qui engendre une insécurité juridique. Dans l'ensemble, les dérogations proposées ne sont pas toutes pertinentes et l'administration demeure la mieux placée pour adapter ses réponses à chaque cas d'espèce.

Permettez-moi, mes chers collègues, de rappeler les nombreuses démarches que le Gouvernement a entreprises depuis le début de ce quinquennat, avec un objectif clair et précis : renforcer l'accessibilité, l'efficacité et la qualité du service rendu, la confiance, la réactivité des services administratifs. Je pense à la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite Essoc, qui consacre et met en oeuvre le droit à l'erreur. Je pense aussi à la simplification des démarches administratives. À titre d'exemple, depuis le début du quinquennat, la part des services publics disponibles en ligne est passée de 63 % 85 % s'agissant des 250 démarches du quotidien. De nombreuses démarches en ligne sont plébiscitées par les Français. Je pense notamment à la réalisation d'une pré-plainte. Cette simplification des démarches administratives est complétée par le programme Services Publics +, qui permet à chaque usager de partager son expérience dans ses relations avec l'administration, de donner son avis après avoir réalisé une démarche en ligne ou de partager de manière plus qualitative une expérience vécue. En un an, ce sont près de 3 millions d'usagers qui ont donné leur avis sur une démarche en ligne. Par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite ASAP, le Gouvernement a également apporté de nombreuses améliorations. Je pense notamment à la dispense de justificatif de domicile pour l'obtention des cartes d'identité, passeports et permis de conduire, avec la généralisation prochaine du dispositif Justif'Adresse. Mes chers collègues, plusieurs chantiers ont été menés pour réformer l'administration dans plusieurs domaines, mais il reste beaucoup à accomplir. Par exemple, Samantha Cazebonne, récemment élue sénatrice des Français de l'étranger, m'a rapporté que ces derniers faisaient face à certaines difficultés pour le renouvellement de leur titre d'identité auprès des services consulaires. C'est un travail de long terme que le Gouvernement a engagé. Il se poursuit avec un objectif : avoir des services publics de proximité plus simples et toujours au service des usagers. La parole

au principe législatif selon lequel le silence gardé par l'administration vaut acceptation de la demande formulée par le citoyen, dans le but, louable, de simplifier son rapport à l'administration.

Aussi, je m'attacherai plutôt à pointer les difficultés liées à l'application du principe selon lequel le silence vaut acceptation et à commenter l'intitulé du texte, qui nous porte vers un sujet au rayonnement bien plus large, puisqu'il s'agit bel et bien d'aborder le rapport des Français à leur administration.

Désormais, le silence gardé par l'administration vaut acceptation. Au fond, il s'agit de deux cas de figure tirant les conséquences d'une lenteur et d'une complexité administratives.

de la réforme de l'État et de la simplification dut réaliser une revue exhaustive des quelque 3 600 procédures prévues par les textes législatifs ou réglementaires et relevant de l'ensemble des ministères : 1 900 procédures seraient encore éligibles à ce dispositif.

Nous le savons, le principe général posé par la loi est affaibli par trop d'exceptions. L'administration elle-même a du mal à s'y retrouver. La crise sanitaire a d'ailleurs éclairé d'une lumière particulière le sujet. Ainsi, la gestion de dossiers communaux par les services de l'État a pu prendre du retard durant les confinements. Selon la direction de l'information légale et administrative, certains d'entre eux, restés lettre morte plus de deux mois d'instruction, se voient rejetés, sans que leur contenu ait été examiné, alors même que le sujet n'entre pas dans les exceptions. Le Gouvernement ne devrait-il pas s'alarmer d'une telle situation ? Le citoyen doit-il souffrir des défaillances de l'administration ? en matière de couacs administratifs vient de nous être donné avec l'affaire de la ferme des mille vaches, portée jusque devant le Conseil d'État. Les juristes y trouveront matière à réflexion, les pragmatiques, un exemple des subtilités paralysantes de notre droit quant à eux, on le devine, incompréhension et sentiment d'injustice. Mettre l'administration au service de l'usager, c'est aussi faciliter l'accès aux services publics,

Alors que la pandémie continue de produire ses effets, la déclinaison sur internet de 250 démarches administratives est annoncée pour 2022. Le Secours populaire et bien d'autres s'inquiètent de cette bascule, qu'ils jugent trop brusque. Elle risque de laisser les personnes fragiles encore un peu plus démunies. La numérisation des services publics en France va-t-elle trop vite ou trop loin ? Elle laisse, en tout cas, trop de monde sur le carreau. Que dire alors du rapport de l'administration avec les usagers ? Que dire encore de cette transition trop souvent mal vécue, qui vide nos territoires ruraux de leurs services publics ? proposition de loi exprime notre volonté de bénéficier d'un système plus efficace, moins compliqué, plus attentif, plus proche du citoyen et, finalement, plus humain. L'administration au service des usagers doit faire preuve de pragmatisme, être l'expression du bon sens. Le couple renforcé préfet-maire, s'il se voyait confier

plus grave encore, de leurs droits.

Nous avons trois fonctions publiques : la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. La crise sanitaire a mis en évidence de nombreuses problématiques majeures,

gouvernement depuis vingt ans à avoir décidé non pas de fermer des services publics, mais de rouvrir 2 000 lieux d'accueil partout en France, pour que les Français, dans chaque canton,

de la Constitution. Nous avons mis en place des dérogations. Nous croyons donc à cette proximité et nous croyons résolument à la déconcentration. Nous ne pouvons pas faire tenir ni tourner notre pays

La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de la proposition de loi initiale.

quelles conséquences tirez-vous du vote massif du Sénat contre la ratification de votre ordonnance sur la réforme de la haute fonction publique ? Je vous ai posé cette question au Sénat, à l'issue d'un débat. Vous n'avez rien répondu. Je suis prêt à tous les dialogues, mais je pense que vous devez répondre à cette question devant notre assemblée, sauf à considérer que notre vote n'a aucune importance

sur l'amendement n° 1. Nous partageons la volonté de l'auteur de la proposition de loi de limiter la marge de manoeuvre laissée au pouvoir réglementaire dans l'aménagement du principe

C'est par des actions opérationnelles, avec les agents publics, sur le terrain, en proximité, que nous donnerons des réponses aux citoyens. C'est pour cela que je me bats et c'est pour cela que les agents publics aujourd'hui innovent et transforment leurs méthodes de travail.

purement et simplement les exceptions réglementaires au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation, nos deux amendements tendent à conserver cette possibilité dans un accompagnement et un encadrement plus précis. Cependant, l'amendement de M. Sueur vise à refondre totalement les exceptions réglementaires prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Or, devant la complexité du droit applicable, nous considérons que cette réforme n'est pas opportune : l'administration, comme le public, y perdrait tout repère.

de manière plus précise et plus détaillée les critères qui devront être respectés par le pouvoir réglementaire pour écarter le principe du SVA. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite voir adopter l'amendement

Comme vous en doutez, je regrette que la commission n'ait pas souhaité donner suite à notre proposition de supprimer purement et simplement l'article L. 231-5, qui ouvre la voie à toutes les dérogations d'ordre réglementaire.

dans le même souci de courtoisie que celui qui vous a fait vous en remettre à notre sagesse, que vous répondiez aux questions qui vous sont posées, sans qu'il soit besoin de durcir le propos pour obtenir enfin une réponse

qui dispose que, « à la demande à l'intéressé [ ...] les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Cet amendement a donc pour objet sa suppression.

nous comprenons l'intention, qui est d'éviter une multiplication de délais différents, nous pensons que l'idée de ce délai unique n'est pas totalement réaliste. Il existe en effet des cas d'urgence qui nécessitent un délai inférieur à deux mois.

Notre idée est que la procédure du silence vaut acceptation doit apporter une réponse aux usagers dans un délai raisonnable. Une procédure de réponse implicite qui serait encadrée par un délai de silence supérieur à six mois n'aurait pas de sens, mais aller jusqu'à six mois préserve la diversité des situations.

L'article 5 prévoit que le délai permettant l'acceptation tacite d'une demande commence, le cas échéant, à courir au moment de sa réception par une administration incompétente, comme c'est actuellement le cas pour les demandes pour lesquelles le silence vaut rejet. Or une telle modification pourrait conduire à une administration à recevoir des demandes pour lesquelles une décision implicite d'acceptation serait déjà acquise en l'absence de toute instruction. En conséquence, cet amendement a pour objet de réécrire l'article 5 afin d'y substituer un nouveau dispositif relatif à la computation des délais

Dans le cadre d'une procédure SVA, une demande de pièces de la part de l'administration n'aurait plus pour conséquence de remettre le compteur à zéro, mais suspendrait simplement le délai qui a déjà commencé à courir à la réception de la demande par l'administration

du délai de recours contentieux. En effet, la suppression de cette condition de forclusion pourrait être particulièrement dommageable pour l'administration, qui s'exposerait à des demandes de motivation tardives.

La commission, dans sa grande sagesse, a choisi de modérer le dispositif de façon pragmatique et réaliste. Je salue de nouveau le travail de Mme le rapporteur, qui a tenu à élaborer un texte équilibré et raisonnable, susceptible de rassembler mes collègues de la commission des lois

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, vous examinez aujourd'hui en nouvelle lecture le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, après avoir constaté mardi en commission mixte paritaire qu'un accord ne pouvait être trouvé. Les deux assemblées ont pourtant considéré, l'une comme l'autre, que la situation sanitaire justifiait de prolonger les outils donnés au Gouvernement pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Les divergences ont principalement porté sur l'échéance à retenir pour la prochaine période de gestion de la crise sanitaire, ainsi que sur les modifications à apporter aux prérogatives accordées au pouvoir réglementaire. Dans la mesure où une motion visant à opposer la question préalable au projet de loi a été déposée, nos débats seront brefs, mais permettez-moi de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce texte, et ce qu'il permet. Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'exprimer devant vous en première lecture, nous n'en avons pas terminé avec l'épidémie de covid. Pour s'en convaincre, il suffit malheureusement d'examiner la situation sanitaire en Europe. À l'heure où je vous parle, nous sommes confrontés à un risque de rebond épidémique, à l'approche de la période hivernale, propice à une accélération de la circulation virale. Pratiquement tous les pays européens font face à une hausse des cas, avec une situation préoccupante en Europe de l'Est. Dans notre pays, on observe depuis plusieurs jours une tendance moins favorable, avec une reprise de la circulation épidémique et, plus récemment, une hausse des hospitalisations et des admissions en soins critiques dans plusieurs territoires. Sans évoquer à ce stade une cinquième vague, nous devons rester vigilants. C'est particulièrement important alors que nous entrons dans une nouvelle période de mise sous tension de notre système de santé par la circulation simultanée de la covid-19 et d'autres maladies saisonnières comme la bronchiolite, la grippe ou la gastro-entérite. Dans les prochains mois, nous devrons donc continuer à lutter contre cette épidémie, en poursuivant toutes les actions nécessaires pour protéger la santé des Français. Ainsi de la vaccination, pour laquelle nous devons convaincre et accompagner nos concitoyens qui ne sont pas encore protégés, en particulier les plus vulnérables. Nous ne devons pas non plus relâcher nos efforts pour la campagne de rappel, qui progresse, mais qui devra progresser encore plus vite. Je m'y emploie avec Olivier Véran. En complément de la vaccination, nous devons conserver la faculté de prendre les mesures de freinage nécessaires pour limiter la circulation du virus. Tel est bien l'objet du présent projet de loi, qui se projette à une échéance adaptée à l'évolution prévisible de l'épidémie. De ce point de vue, le choix du 31 juillet prochain est pertinent. Nous savons très bien dès à présent qu'il nous faudra vivre avec le virus au moins jusqu'à l'été, et la période hivernale amplifiera sa circulation dans les prochains mois. Je rappelle en outre que la date du 31 juillet a été soumise respectivement au conseil scientifique et au Conseil d'État, qui ont pleinement validé cette orientation, chacun dans son office. Cette prorogation avait comme corollaire un renforcement de l'information du Parlement. Le rapport d'étape qui sera remis par le Gouvernement d'ici la mi-février permettra ainsi de disposer d'une clause de revoyure, qui pourra bien entendu donner lieu à un débat en commission ou en séance, en présence du Gouvernement. La remise d'un second rapport d'ici la mi-mai et la production de synthèses mensuelles sur les mesures prises et leur impact sur la situation sanitaire compléteront l'ensemble des initiatives déjà prises par ailleurs pour assurer une information pleine et entière du Parlement. Quant aux outils de gestion de l'épidémie, le projet de loi permet de les conforter et de les améliorer sur la base du retour d'expérience acquis ces derniers mois, sans en bouleverser l'économie générale. Il permettra ainsi de mieux contrôler le respect de l'obligation vaccinale pour les publics concernés, de lutter avec davantage de rigueur contre les fraudes au passe sanitaire, et de renforcer la campagne de dépistage et de vaccination dans les établissements scolaires. Les modalités de recours au passe sanitaire ont par ailleurs été précisées, en prévoyant que sa mise en oeuvre sera justifiée par la circulation virale ou ses conséquences sur le système de santé, selon des indicateurs que le pouvoir réglementaire devra prendre en compte. Sans imposer une logique de territorialisation du passe selon un critère sanitaire unique et une valeur de référence directement fixée dans la loi, ces précisions réaffirment le principe d'une mise en oeuvre du passe strictement adaptée et proportionnée aux risques sanitaires encourus. Comme le Gouvernement l'a déjà indiqué, l'application du passe sanitaire tel que nous le connaissons depuis l'été sera réexaminée dans les prochaines semaines, et ajustée si la situation le justifie. Le projet de loi comprend enfin un nombre ciblé de mesures d'accompagnement, qui permettront de faire face aux conséquences de la crise sanitaire, en matière d'activité partielle, de fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales ou de durée de validité de certaines décisions administratives. Malgré l'absence d'accord entre les deux assemblées, le projet de loi qui vous a été transmis reprend plusieurs dispositions importantes adoptées par le Sénat en première lecture. Je pense en particulier à la Je pense en particulier à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en Martinique, adoptée en concertation avec votre commission des lois. La situation dans ce territoire le justifie pleinement, avec une circulation virale qui se maintient à un niveau élevé, un taux d'occupation des lits de réanimation supérieur à 100 % et une couverture vaccinale encore insuffisante. Je pense également aux dispositions précisant le périmètre de l'obligation vaccinale dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, insérées sur l'initiative de Mme Gruny, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Elles permettront de sécuriser juridiquement les orientations retenues depuis le mois d'août pour tenir compte des spécificités de ce secteur. Je Je pense enfin à l'article permettant d'accompagner la création de systèmes d'information analogues à SI-DEP en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. C'était une demande forte des élus de ces territoires, et je me félicite que nous puissions directement y répondre dans ce projet de loi pour renforcer localement la gestion et le suivi de l'épidémie. Enrichi par ces compléments, le projet de loi qui vous a été transmis est un texte équilibré et adapté à la situation sanitaire des prochains mois. Les prérogatives qu'il permettra de mobiliser s'inscrivent en effet dans un régime juridique précis et exigeant, qui a pleinement fait ses preuves pour concilier l'objectif de protection de la santé publique avec le respect des droits et libertés. Le Sénat a d'ailleurs largement contribué à définir et à préciser ce cadre d'action lors des différents rendez-vous législatifs que nous avons eus depuis mars 2020. Les différentes mesures prises en application de ce régime devront toujours répondre aux exigences essentielles de nécessité et de proportionnalité, dont le respect sera placé sous le contrôle du juge administratif, y compris par des procédures de référé d'urgence. J'ajoute également que, si le Gouvernement était amené, compte tenu de la situation sanitaire, à déclarer à nouveau l'état d'urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire national, le Parlement devrait être impérativement saisi pour autoriser sa mise en oeuvre au-delà d'un mois. Encore heureux ! Vous l'aurez compris, ce projet de loi, à l'image des précédents, permettra de protéger la santé des Français en limitant au mieux l'impact des mesures prises sur leur vie quotidienne. C'est un équilibre difficile, sans cesse renouvelé face à l'évolution de la circulation du virus, à l'irruption de nouveaux variants et à l'état des connaissances. Cet équilibre, le Gouvernement s'emploie chaque jour à le maintenir et à anticiper, car gouverner, c'est prévoir. Le projet de loi permettra de poursuivre dans cette voie, en disposant des moyens nécessaires pour gérer la suite de la crise sanitaire, avec toutes les garanties requises en termes de libertés publiques. Permettez-moi de conclure en rappelant que le désaccord entre les deux assemblées sur ce texte n'ôte rien à l'importante mobilisation du Parlement depuis le début de la gestion de cette crise. À cet égard, permettez-moi de saluer une fois encore la participation du Sénat à chacun des rendez-vous législatifs que nous avons eus depuis bientôt deux ans sur ce sujet, souvent dans des conditions de travail difficiles, imposées par les circonstances. Le Gouvernement restera fidèle à l'approche retenue depuis le début de la crise, en prenant les mesures nécessaires et proportionnées à l'évolution de la situation pour protéger la santé de nos concitoyens dans les meilleures conditions. Je ne doute pas que le Sénat restera fidèle à la sienne, en portant un regard sévère,

Madame la présidente,

au début de l'année 2020, notre pays s'est trouvé pris au dépourvu : pas de masques, pas de tests de dépistage, pas de gel hydroalcoolique, pas de pratique des gestes barrières, pas de pratique massive du télétravail, pas de médicaments, pas de vaccins. notre pays n'a été logé ni à pire ni à meilleure enseigne que beaucoup d'autres. Sauf peut-être, en ce qui concerne la disponibilité des masques et des tests de dépistage

l'ensemble de ces dispositifs concrets et pratiques, aussi bien d'ordre médical que relevant de l'organisation de la société, ne pouvaient être mis en oeuvre qu'il a fallu procéder d'une autre manière pour enrayer l'épidémie. Ce fut le premier confinement madame la ministre, le Sénat a répondu présent. Il l'a fait sans porter de jugement sur les responsabilités de la situation à laquelle nous étions confrontés, mais parce qu'il lui est apparu alors que c'était le seul moyen de se donner une chance de limiter la propagation d'une épidémie qui saturait déjà les services hospitaliers et, en particulier, les services de réanimation. Cette épidémie a connu de nombreux rebondissements. L'expérience acquise depuis mars 2020 doit nous conduire à considérer aujourd'hui que la restriction des libertés individuelles n'est ni le moyen unique ni même le moyen principal qu'il faut mettre en oeuvre pour juguler l'épidémie. La situation est tout de même bien différente, sur tous les points que je viens d'évoquer, par rapport à ce qu'elle était il y a dix-huit mois. Même

il y a seulement quelques mois. Non seulement le Sénat de la République a accepté, en mars 2020, en contradiction avec ce qui fait son identité profonde, des restrictions inévitables à nos libertés, mais il a continué à accorder au Gouvernement, chaque fois qu'il les lui demandait, les moyens d'action qui lui paraissaient proportionnés- après l'avoir vérifié, bien sûr -à la situation sanitaire qu'il s'agissait de maîtriser du mieux que l'exécutif pouvait le faire, avec l'aval du Parlement. Il l'a fait, encore, quand il s'est agi d'imposer l'utilisation du passe sanitaire à l'entrée des cafés, restaurants, salles de spectacles et lieux rassemblant de nombreux concitoyens, tels les foires, marchés et salons. On ne pourra pas dire que le Sénat n'a pas répondu présent. On ne pourra pas dire que le Sénat n'a pas assumé ses responsabilités. Toutefois, pour notre assemblée, la contrepartie de cet engagement aux côtés des autorités sanitaires, c'est l'exigence d'un contrôle parlementaire qui permet d'adapter, pas à pas, les instruments de la lutte contre le covid-19 à la réalité de la situation sanitaire. Si le régime de l'état d'urgence sanitaire est un régime temporaire qui, dans l'esprit du législateur, peut être activé à tout moment en fonction de l'évolution de l'épidémie,

Madame la ministre, aujourd'hui encore, le Sénat ne s'oppose pas à ce que les instruments de la lutte contre l'épidémie soient prolongés. Mais de la même façon qu'il l'a toujours fait, il veut que ce soit sous son contrôle et sous le contrôle de l'Assemblée nationale. Ces droits du Parlement, nous ne pouvons les laisser prescrire, pour une raison très simple, c'est qu'ils ne nous appartiennent pas.

prises. Je dois vous dire, madame la ministre, à la fois ma tristesse et mon étonnement de voir que ce que le Gouvernement a accepté, par exemple il y a trois mois et demi bientôt pour la durée de vie du passe sanitaire, il le refuse pour les mois à venir. Qu'est-ce qui a donc changé dans les déterminants de la position du Gouvernement ? Je ne parviens pas à croire

À la tristesse s'ajoutent donc l'incompréhension et le mécontentement face au non-respect de principes fondamentaux de nos institutions démocratiques. C'est la raison

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la crise est toujours là et la menace d'une nouvelle vague de l'épidémie se fait sentir. Nous l'avons dit et répété, et nous le ferons encore et toujours, malgré la lassitude qui pourrait nous gagner : l'urgence n'est plus là. Rien ne peut plus justifier aujourd'hui la perpétuation d'un état d'exception qui met à l'écart le Parlement et porte atteinte, dans un même mouvement, à des libertés essentielles de nos concitoyens. par exemple, le nouveau rôle dévolu aux directeurs d'école, désormais habilités à exercer une forme de police sanitaire ? Nous l'avons dit et répété, la conviction démocratique devrait exiger que le Parlement décide et que le Parlement prenne le temps de décider. Prenons ce débat. Pourquoi une telle précipitation ? Madame la ministre, la France n'est plus à l'arrêt, l'épidémie a reculé grâce à la vaccination, même si la vigilance doit rester de mise. Pourquoi, dans ces

le Parlement doit reprendre le pouvoir. Les assemblées peuvent être saisies à tout instant, de nuit comme de jour, y compris pendant l'interruption des travaux liée aux prochains scrutins électoraux, pour débattre, proposer, La gestion solitaire de la crise sanitaire par Emmanuel Macron n'est plus acceptable. Il ne faut pas s'habituer à ces conseils de défense opaques, dépourvus de fondement constitutionnel, où les décisions sanitaires se prennent. Dois-je rappeler, une fois encore, que la santé ne fait pas partie du domaine réservé du Président de la République ? Il revient maintenant au Parlement de décider, par la loi, de chaque étape de l'action sanitaire, de manière régulière. et la santé de notre peuple ne doivent plus être une affaire de décret ou d'ordonnance, mais bien une affaire reprise en main par ses représentants, par la démocratie. La question de l'hôpital public est à ce titre symbolique. Le Gouvernement nous promène dans les méandres du passe sanitaire, de cette société de vigilance chère au Président de la République, alors que, dans le même temps, l'hôpital public connaît une crise sans précédent, faisant courir le risque d'un effondrement de notre système de santé en cas de nouvelle vague. Oui, le Gouvernement fait courir de graves risques à notre pays en ne prenant pas les mesures d'urgence. Or là, il y a urgence, pour redresser l'hôpital public et rouvrir, ici et maintenant, les milliers de lits

notre part, alerté sur le danger d'essayer d'aménager un dispositif de restriction des libertés aussi fort que cet état d'urgence et son excroissance, le passe sanitaire.

améliorait fortement le dispositif gouvernemental, mais il ne s'opposait pas frontalement à la logique autoritaire et infantilisante qui est celle du Gouvernement. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE se prononcent clairement contre la prorogation de l'état d'urgence et du passe sanitaire. Ils rappellent que les nécessités de l'heure sont le redressement de l'hôpital public, la prise en compte du devenir des personnels souvent démissionnaires ou suspendus du fait de la non-vaccination, mais certainement pas cette captation du pouvoir par l'exécutif, qui accélère le passage

la question préalable qui sera proposée par notre commission des lois. Quelques mots enfin, madame la ministre, pour vous dire que j'attends avec gourmandise la décision éventuelle du Conseil constitutionnel

il y a des commissions mixtes paritaires qui, lorsqu'elles échouent, nourrissent de profonds regrets. Mon groupe s'était prononcé majoritairement contre ce projet de loi, y compris dans sa version sénatoriale, et cette commission Bien sûr, nous avions vu l'effort du Sénat visant à ramener la fin des dispositifs exceptionnels à la date du 28 février 2022. Certains de mes collègues avaient d'ailleurs déposé des amendements en commission, afin que la date choisie soit celle du 15 février. Nous avions vu également le travail fastidieux de notre hémicycle au sujet de l'encadrement du passe sanitaire. La territorialisation du dispositif était le minimum attendu. Seulement, même en l'état, le projet de loi resterait encore peu satisfaisant à mes yeux. Aussi, vous imaginez bien que ce nouveau texte, qui reprend l'essentiel des positions initiales de l'Assemblée nationale, n'arrange rien. D'abord, le choix de la date représente un obstacle presque insurmontable. Il va de soi que j'entends les arguments du Gouvernement en faveur du 31 juillet 2022 dans la gestion de cette crise : simplicité, efficacité, performance, optimisation. Tout le champ sémantique de la modernité managériale pourrait s'y trouver associé. Pourquoi alors s'embarrasser de vieux outils, ceux du contrôle parlementaire et de l'équilibre institutionnel ? Il ne faut cependant pas s'y tromper, l'État n'est pas une entreprise, et le Parlement n'a pas à externaliser ses compétences au profit d'autres conseils, sans doute érudits, mais dépourvus de toute légitimité démocratique. cette légitimité n'est pas encore tombée en désuétude ! Aussi, je crois que c'est à tort que sera retenue la date du 31 juillet 2022. Bien entendu, le chemin choisi par le Sénat était le bon, avec l'avancement de la date au 28 février pour la fin des dispositifs, mais il m'est apparu encore insuffisant. Il ne s'agit pas de nier la situation sanitaire ni de critiquer aveuglément la gestion de la crise. Toutefois, face à ces régimes d'exception qui perdurent, il faut savoir garder un cap. Le nôtre a toujours été le même : tout état d'exception ne peut être envisagé que comme une mesure provisoire et extraordinaire. Il ne saurait nullement s'installer comme un paradigme normal de gouvernement. Or c'est ce qui est en train d'advenir avec ce projet de loi. Ensuite, il y a ce très controversé passe sanitaire, qui devait demeurer un dispositif exceptionnel en vue d'inciter nos concitoyens à se vacciner. Je n'y étais déjà pas favorable en juillet dernier, mais force est d'admettre qu'il a pu contribuer à éviter un rebond épidémique estival. Mais alors, pourquoi ne pas profiter du succès du dispositif pour y mettre fin ? La population française est désormais largement vaccinée, et nous ne sommes plus à la traîne comme on pouvait l'entendre voilà encore quelques mois. Pourquoi donc maintenir ce dispositif si attentatoire aux libertés individuelles ? Pourquoi vouloir pérenniser un outil source d'incompréhension et de frustration ? Faut-il encore le rappeler, en matière de libertés publiques, la liberté est la règle et la mesure de police doit à tout prix demeurer l'exception. Nous avons su, en responsabilité, admettre l'exception pour un temps, mais revenons désormais au principe : celui de la liberté, qui fait l'essence de notre nation Enfin, il y a la question de l'accès aux données virologiques des élèves dans les établissements scolaires. Nous y sommes farouchement opposés. Là également, il faut trouver d'autres moyens. La position du Sénat était la bonne à mes yeux. Il reste, pour conclure, que nous aurions aimé qu'un débat puisse de nouveau avoir lieu sur ces sujets si graves afin que chacun ait la possibilité de réaffirmer ses positions. Le groupe du RDSE, fidèle à son habitude, se prononcera donc contre la motion déposée. La parole

le Gouvernement, insensible aux arguments du Sénat et au mécontentement croissant de la population, n'a pas infléchi sa position à l'égard de sa stratégie de sortie de crise. Il fait le choix, encore, de l'autorité et de la concentration du pouvoir au détriment de notre bon fonctionnement démocratique, de nos libertés et de la préservation du secret médical. J'ai déjà exprimé ici ma ferme opposition aux dispositifs proposés dans ce projet de loi. Je réaffirme ce désaccord. Tout porte à penser que ce virus ne disparaîtra pas totalement de nos vies. Le Gouvernement nous condamne-t-il donc à vivre sous le joug d'infinies prorogations l'état d'urgence en espérant une éventuelle disparition du virus ? Ce risque, je refuse de l'accepter. Le seul choix possible est d'apprendre à vivre avec le virus. Il nous faut pour cela mettre en place des solutions pérennes qui nous permettront de sortir du cercle vicieux des prorogations successives d'états d'exception. Vivre avec le virus implique de posséder un système hospitalier fonctionnel. Or le conseil scientifique estime que 20 % des lits d'hôpitaux sont actuellement indisponibles. Les personnels soignants sont exténués, au bord de la rupture. Les chiffres relatifs à l'absentéisme et aux nombreux départs le prouvent. Cette situation est la conséquence directe directe de la politique de santé menée par le Gouvernement, qui est inefficace. Vivre avec le virus, c'est aussi optimiser l'utilisation des armes que nous possédons. Le vaccin a fait ses preuves. Pourtant, certains de nos concitoyens sont toujours réticents à son utilisation. D'autres, souvent précaires, sont exclus du système de vaccination. La pédagogie envers ces publics doit être développée, sur la possibilité de recourir à une troisième dose de vaccin. J'appelle aussi le Gouvernement à agir pour faire lever les brevets sur les vaccins.

pourtant la motion, cette issue étant la seule envisageable face à un gouvernement qui persiste à refuser la tenue d'un débat digne de ce nom. La parole

que l'Assemblée nationale s'apprête à conférer à votre gouvernement, madame la ministre, sans qu'il y ait de contrôle parlementaire possible pendant cette période. Nous ne pouvons pas accepter que l'Assemblée nationale nous renvoie un texte qui organise l'abandon de ses propres missions constitutionnelles de contrôle de l'action du Gouvernement pendant de nombreux mois, alors qu'un certain nombre de mesures restreignent les libertés.

le Parlement dans le congélateur pendant neuf mois, c'est affaiblir la lutte contre la crise sanitaire. Or ce n'est pas le moment, car, vous l'avez indiqué, les chiffres, à l'est de l'Europe en particulier, montrent que rien n'est terminé. Ils montrent aussi que, là où la vaccination est questionnée, les contaminations galopent et multiplient les risques de mutation. Rien n'est donc gagné et rien ne saurait être mis en pilotage automatique.

les procurations pour les prochaines élections, le 5 décembre 2021, à l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous considérons enfin que, sans définition sur ce que sera, dans quelques semaines, un parcours vaccinal complet, tout cela est prématuré.

Pour toutes ces raisons, madame la ministre, parce que nous n'avons pas aujourd'hui de réponses du Gouvernement sur ces sujets, nous ne pouvons pas accepter les propositions qui viennent de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons pouvoir continuer le débat sur ce texte, sur la base de nos principes et de nos inquiétudes. La parole

l'échec de la commission mixte paritaire a mis en exergue les profondes divergences entre les textes issus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le vote émis hier soir par nos collègues députés ne pouvait que confirmer les désaccords entre nos deux chambres.

Quelques réserves sur ce dernier point : l'intérêt du passe sanitaire a été compris par les Français, mais, malheureusement, ils sont encore trop nombreux à ne pas être vaccinés. Le virus circule entre les départements. Les connaissances sur l'épidémie sont évolutives et l'apparition d'un nouveau variant encore plus contagieux reste une hypothèse crédible. Une circulation accrue du virus au cours de la période hivernale n'est plus une probabilité. (OMS) elle-même s'alarme aujourd'hui du rythme « très préoccupant » de la transmission du virus en Europe. L'efficacité de la protection du vaccin semble baisser au cours du temps, d'où l'importance de la campagne de rappel. Le variant delta, identifié désormais dans 100 % des séquences analysées, présente une contagiosité plus élevée. « Nous n'avons pas atteint le seuil d'immunité collective », selon le Conseil d'État et l'OMS. Comment imaginer que le texte dénaturé qui est sorti de notre assemblée après la première lecture, avec l'assouplissement des mesures qu'il aurait engendré, aurait pu répondre à une nouvelle vague déjà forte à nos frontières et perceptible en France ? Dire que la volonté du Gouvernement était de dessaisir le Parlement de ses prérogatives ou encore qu'il voulait enjamber les élections à venir est, de la part de la majorité des membres du Sénat, une figure de style. ! Nous le savons tous ici : en cas de réenclenchement du régime de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement fera toujours appel à la validation du Parlement au bout de quatre semaines pour les mesures les plus lourdes. Enfin, comment peut-on limiter ce débat à une problématique franco-française ? En Europe, les hospitalisations liées au covid-19 ont plus que doublé en une semaine. Le nombre de nouveaux cas par jour est en hausse depuis près de six semaines. Le nombre de nouveaux morts par jour est lui aussi en hausse depuis un peu plus de sept semaines, avec environ 250 000 cas et 3 600 décès quotidiens. Et nous aurions dû baisser la garde ? Le personnel soignant, sur le pont depuis l'origine de cette crise, n'aurait pas supporté le changement de cap que vous proposiez à l'aube de la période hivernale. L'expérience acquise depuis dix-huit mois doit nous conforter dans l'utilisation d'une méthodologie et d'outils éprouvés et compris par l'ensemble de nos concitoyens. Le « en même temps », qui allie sécurité sanitaire et liberté individuelle, a largement fait ses preuves et continue à les faire. Le contretemps que proposait le Sénat en modifiant toute l'architecture du système mettait, quant à lui, en péril les bons résultats déjà obtenus et, surtout, fragilisait la protection que nous devons à nos concitoyens. Aussi, je me réjouis du vote des députés hier soir. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, mais aussi parce que nous avons toujours été contre les débats tronqués, nous nous opposerons à la motion qui sera proposée tout à l'heure. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que le temps presse, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à s'accorder sur un texte commun. Il nous faut cependant décider des moyens dont le Gouvernement pourra disposer afin de gérer la pandémie en cours. Bien sûr, la situation est bien meilleure qu'il y a quelques mois. Les Français ont fait maintes fois la preuve de leur sens des responsabilités en respectant, depuis plus d'une année maintenant, les mesures barrières. Ils ont également largement plébiscité la vaccination, avant même que le passe sanitaire ne les y incite plus fortement. L'amélioration de la situation sanitaire dans notre pays, qui compte parmi les mieux vaccinés au monde, ne doit pas nous faire baisser la garde : la pandémie est toujours en cours.

Plus près de nous, plusieurs pays européens connaissent une reprise épidémique qui nous appelle à rester vigilants. Près de 40 000 contaminations quotidiennes ont ainsi été recensées au Royaume-Uni sur les sept derniers jours. L'Allemagne a vu les hospitalisations liées à la covid-19 grimper de 40 % en une semaine. Nos propres services de santé enregistrent déjà une hausse des hospitalisations, même si la vaccination permet à notre pays de mieux résister. En effet, le vaccin réduit de 92 % le risque d'hospitalisation chez les plus de 50 ans. nous devons maintenir notre vigilance dans les prochains mois. Le projet de loi que nous examinons de nouveau aujourd'hui détaille les mesures dont l'exécutif estime avoir besoin pour faire face à la crise. Le passe sanitaire, et c'est normal, concentre toutes les attentions. Sa mise en place ayant permis d'accélérer significativement le taux de vaccination de la population, certains souhaitent le voir disparaître en considérant qu'il a rempli sa mission. Nous savons cependant que les anticorps contre la covid-19 ne sont pas éternels. Une troisième dose sera sans doute nécessaire. Si tel est le cas et que nous ne souhaitons pas recourir à la vaccination obligatoire, il faudra sans doute maintenir le passe Reste la délicate question de la durée des pouvoirs consentis au Gouvernement. C'est sur ce point que porte le plus grand désaccord. Le Sénat aurait voulu un nouveau débat à la fin du mois de février prochain, juste avant la suspension des travaux parlementaires. Le Gouvernement et les députés souhaitent, quant à eux, que les mesures envisagées durent jusqu'à la fin du mois de juillet prochain, c'est-à-dire lorsque le Président de la République aura été élu et le gouvernement formé. Lors des prochains mois, la gestion de la crise sanitaire devra s'accommoder de la campagne pour l'élection présidentielle. Si la situation l'exige, le Parlement peut effectivement siéger durant la suspension de ses travaux, mais le contexte de la campagne n'offre pas nécessairement les meilleures conditions pour la tenue sereine d'un tel débat. Il n'en reste pas moins que les pouvoirs en cause sont exceptionnels, et qu'il est délicat de les confier à l'exécutif jusqu'à la fin juillet- un exécutif que nul ne connaît encore, Il n'y a pas de réponses simples à toutes ces questions. Beaucoup de doutes planent sur les prochains mois, mais nous avons néanmoins une certitude : la pandémie ne va pas disparaître immédiatement, et notre pays, comme le reste du monde, va devoir continuer à lutter contre le virus. La parole

soumet le Gouvernement, nous nous retrouvons pour une nouvelle lecture de ce texte. Que de regrets ! Que d'amertume ! Le Sénat, une fois encore, avait fait preuve en première lecture réel esprit de responsabilité, notamment au travers du travail remarquable de son rapporteur, Philippe Bas, dont la logique constructive et rationnelle a été animée par une même exigence depuis le début de la crise

entre la préservation de la santé des Français et le respect des principes de l'État de droit, d'une part ; entre un régime d'exception portant en lui-même des moyens exceptionnels de gestion de crise et les libertés fondamentales inscrites dans notre Constitution,

L'Assemblée nationale a choisi de rétablir largement son texte initial, en particulier sur ses mesures centrales : la prorogation jusqu'au 31 juillet de la plupart des régimes dérogatoires et mesures afférentes, y compris le passe sanitaire, l'absence de territorialisation de son application, ou encore l'accès des directeurs d'établissements scolaires aux données virologiques de leurs élèves ; voilà, pour nous, autant de lignes rouges franchies. L'argument du rapporteur de l'Assemblée nationale suivant lequel la sortie des régimes actuels d'urgence sanitaire serait source d'instabilité et d'imprévisibilité apparaît quelque peu douteux. En effet, les mesures proposées par le Sénat, au travers de deux nouveaux dispositifs, comprenaient pour l'essentiel des outils déjà existants, sous des formes et des modalités adaptées à la situation sanitaire actuelle. Le texte voté la semaine dernière par notre assemblée prévoyait ainsi de maintenir à la disposition du Gouvernement des pouvoirs exceptionnels de régulation des déplacements et des rassemblements, ou encore de mise en oeuvre du passe sanitaire. En contrepartie, il fixait un rendez-vous parlementaire en février prochain, afin d'amener l'exécutif à rendre compte formellement devant le Parlement de son usage de ces pouvoirs, mais aussi afin d'évaluer la proportionnalité des mesures exceptionnelles à l'aune de l'évolution de la situation épidémique. Aucun argument sérieux ne nous a été opposé sur la question de la date de fin du dispositif sanitaire, date qui n'est qu'un nouveau rendez-vous

de la Constitution ou remise de rapports -ne sauraient nullement remplacer la discussion en bonne et due forme d'un projet de loi aux termes duquel le Parlement autorise le Gouvernement à continuer d'assumer ses pouvoirs. nationale un nouvel affaissement de la mission législative du Parlement, une volonté affichée de s'affranchir de sa mission de contrôle, sous prétexte que la gestion de crise exige une prise de décision rapide.

le rapporteur l'a rappelé, en mars 2020, nous étions démunis : pas de masques, pas de tests, pas de gel hydroalcoolique, pas de vaccin, pas de traitement ! Aujourd'hui, nous avons progressé dans tous ces domaines, y compris sur la connaissance même du virus. Alors, est-il légitime de réduire ainsi le contrôle parlementaire exercé sur des pouvoirs dérogatoires accordés à l'exécutif, sous prétexte de l'approche de grandes échéances électorales ?

Enfin, la disposition permettant aux directeurs d'école de prendre connaissance du statut virologique des élèves semble véritablement porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Face à l'opposition intransigeante du Gouvernement et de sa majorité, notre rapporteur nous invite à maintenir notre position historique et nous proposera tout à l'heure d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable. Convaincus du fait que nous ne pouvons pas vivre indéfiniment dans un régime d'exception et fermement opposés à la méthode disproportionnée employée par le Gouvernement, les élus de notre groupe voteront cette motion.

la réticence des deux tiers des parlementaires à vous laisser les mains libres pendant huit mois, malgré le mauvais signal envoyé d'un désir tout politique d'enjamber la consultation légitime du Parlement en cas de reprise épidémique à une période peut être trop proche des échéances électorales aux yeux du président,

sanitaire en tant que tel, c'est-à-dire son simple pouvoir de limiter l'accès des personnes non vaccinées ou non testées à certains lieux de vie a été très peu étudiée et encore moins quantifiée sur le moyen terme. Ces derniers mois, il nous est apparu que son efficacité était surtout liée à l'incitation à la vaccination qu'il a suscitée ; notre groupe reconnaît à cet égard la force de l'outil vaccinal dans la lutte contre la pandémie. parle de mettre en place des mesures restrictives pour lutter contre le virus, un déploiement efficace de l'outil vaccinal. Les plus fragiles, les plus précaires, les plus éloignés de l'épicentre de notre vie sociale ne sont pas suffisamment vaccinés. Le passe sanitaire aura-t-il un effet protecteur sur ces populations ? À ce jour, moins de la moitié des personnes éligibles à la troisième dose, c'est-à-dire les plus vulnérables, celles qui en ont particulièrement besoin, y ont eu recours. vous avez depuis le début des débats refusé de parler de la troisième dose, de son intégration éventuelle au passe sanitaire, de sa généralisation et même de l'échec de la campagne actuelle pour le public cible. La moitié des personnes complètement vaccinées aujourd'hui ont reçu leurs deux doses avant le 1 juillet 2021. Comment pouvez-vous présenter un texte permettant des mesures extraordinaires jusqu'en juillet 2022 sans discuter de cette baisse annoncée de l'immunité de la population générale vaccinée ?

Pour l'instant, non : ce rappel vaccinal n'est pas encore en population générale ». Pourquoi ne voulez-vous pas en discuter maintenant ? Pourquoi ne répondez-vous jamais aux questions qui vous sont posées par les parlementaires du Sénat, madame la ministre ?

faible. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

la fin de non-recevoir qu'il a opposée à nos amendements, que nous estimions pourtant constructifs et raisonnables, nous ont laissé sans espoir de parvenir à vous convaincre de faire encore évoluer le texte après l'échec de la commission mixte paritaire. Le travail parlementaire ne peut ressembler à une sorte de théâtre d'ombres. Nous n'allons donc pas faire semblant, ce soir, de penser qu'il y a encore une chance que vous accédiez à nos raisons. Évidemment, ce ne sont que nos raisons ; il faut il faut que nous ayons, nous aussi, l'humilité d'admettre que d'autres points de vue que le nôtre peuvent être entendus. Mais pour qu'ils le soient, encore faudrait-il que l'on perçoive

prolonger un passe sanitaire créé pour trois mois et demi jusqu'en juillet de l'année prochaine, c'est-à-dire pour encore huit mois et demi. Bien sûr, rien ne vous impose d'utiliser ce passe sanitaire. D'ailleurs, le comité scientifique vous a recommandé de préparer la sortie de ce dispositif. Il a raison : nous l'avons pris au mot et nous avons organisé cette sortie. Je suis

où l'immunisation de la population par le vaccin n'est pas suffisante, tout en délivrant de cette contrainte les habitants des territoires qui ont été massivement vaccinés.

sans avoir accepté la proposition du Sénat et de votre propre initiative, j'y verrais naturellement une reconnaissance de la qualité de notre travail, mais j'aurais préféré que cette reconnaissance s'exprime au moment du vote de la loi

que vous nous l'avez demandé. Mais aujourd'hui, ce que vous demandez à l'Assemblée nationale, car nous refusons de le faire, c'est d'offrir au Président de la République qui

-qui montrent que la manière dont nous devons affronter cette épidémie a profondément changé de nature. Ce n'est pas aux Français vaccinés qu'il faut aujourd'hui demander la protection des réfractaires derniers d'assurer eux-mêmes leur propre protection, car ils ont eu, grâce à notre travail collectif, tous les moyens de se protéger et ils les ont toujours.

contre le covid-19, tout en nous réservant la possibilité, jusqu'au 28 février prochain, de prendre des mesures plus énergiques si nous ne pouvions pas affronter l'épidémie autrement.

aux chefs d'établissement scolaire de procéder à des discriminations entre les élèves en fonction de leur statut viral ou vaccinal.

en fonction de la décision de leurs parents de les faire vacciner ou non. S'il s'agissait seulement de faciliter les campagnes de vaccination, les chefs d'établissements n'auraient nul besoin d'accéder aux informations médicales relatives

avec son médecin, son laboratoire d'analyses biologiques, la plateforme de l'assurance maladie, puis de s'isoler, de respecter un certain nombre de recommandations qui lui sont faites, mais l'employeur n'est pas saisi. De la même façon, un élève

nous ne pouvons que rejeter les propositions que vous nous faites, non sans avoir essayé de les amender pour parvenir à un texte qui, je le pense, aurait

attaché au rôle du Parlement, mais de refuser que le Sénat puisse jouer son rôle en nouvelle lecture. nouvelle lecture. Il ne faut pas céder à la désespérance. La base de la pédagogie, c'est la répétition. L'Assemblée nationale refuse notre texte. La Constitution nous donne la possibilité de le proposer de nouveau. Pourquoi

Le Sénat a assumé ses responsabilités pour faire face à l'épidémie qui sévit depuis bientôt deux ans. Nous ne nous sommes jamais dérobés, madame la ministre, lorsqu'il a fallu avaliser ou proposer des mesures, y compris lorsqu'elles étaient difficiles, pour gérer cette crise, mais notre groupe pense qu'il est désormais de son devoir de dire « stop » au mode de fonctionnement du Gouvernement. Vous connaissez la position majoritaire des parlementaires, madame la ministre, mais vous n'en tenez aucun compte.

comme pour d'autres textes que nous avons examinés sur d'autres sujets, nous avons toujours l'impression, au Sénat, d'argumenter face à un mur et, finalement, de ne jamais être entendus.

Le scrutin est ouvert.